chacune et chacun à veiller au respect des distances de sécurité. Je rappelle que tous les orateurs, y compris les membres du Gouvernement, s'exprimeront depuis leur place, sans monter à la tribune. Dans la discussion générale, la parole est à M. Pascal Savoldelli, auteur de la proposition de loi. Monsieur

Ces travailleurs se sont d'ailleurs trouvés en première ligne durant la crise épidémique du Covid-19, bien malgré eux, en plein confinement, alors que leur activité n'était pas toujours essentielle, parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Ce sont les chauffeurs de VTC, les coursiers, ou encore les livreurs, tous au service de plateformes numériques de travail, ceux que l'on nomme couramment « travailleurs ubérisés Il s'agit d'un enjeu d'actualité particulièrement important. Je tiens à remercier mes collègues Michel Forissier, Catherine Fournier et Frédérique Puissat, ainsi que la commission des affaires sociales, de leur rapport d'information portant sur le droit social applicable aux « travailleurs indépendants et économiquement dépendants » ; ce rapport fort intéressant démontre l'importance et l'actualité de ce sujet qui pourrait, peut-être, nous rassembler au-delà de nos différences politiques. Notre proposition de loi tend à offrir un statut protecteur aux travailleurs des plateformes numériques. Cela dit- c'est assez rare pour qu'on le souligne -, ce texte est le fruit d'un travail collectif de plus de deux ans.

des travailleurs des plateformes, mais aussi des acteurs syndicaux, universitaires et politiques. La proposition de loi que nous vous présentons aujourd'hui est donc le fruit d'un véritable travail collectif, concerté, singulier par sa diversité et directement lié aux réalités de terrain. Elle traduit par conséquent des volontés exprimées par les travailleurs des plateformes eux-mêmes.

Nous avons également discuté avec des travailleurs qui se sont organisés et ont pris des initiatives locales, plus éthiques et protectrices, pour proposer des alternatives concrètes à ces géants du numérique : je pense notamment à CoopCycle, une fédération de coopératives de coursiers à vélo.

nous ont aussi fait part de l'emprise économique que peuvent exercer ces géants du numérique sur les commerces locaux. L'arrivée sur le marché de ces plateformes peut certes paraître bénéfique, au départ, pour certains commerces. Toutefois, peu à peu, la part accordée aux plateformes gagne du terrain

Nous sommes face à une stratégie classique visant à casser le marché pour le conquérir et aboutir, à terme, à une situation de monopole par des pratiques de dumping social. Nous proposons donc, par le biais de cette proposition de loi, de renforcer les droits des travailleurs et de renvoyer ces entreprises du numérique à leurs responsabilités à l'égard de plusieurs aspects. nous entendons intégrer le statut de ces travailleurs à la septième partie du code du travail, afin de leur offrir un contrat de travail véritablement protecteur et assimilé au salariat. Cette forme de salariat autonome devrait permettre de leur assurer la sécurité dont ils ont besoin tout en préservant l'autonomie qu'ils ont dans l'organisation de leur travail. Ensuite, nous proposons d'organiser leur accès à une véritable protection sociale : aujourd'hui, il suffit qu'un de ces travailleurs tombe malade ou ait un accident du travail pour qu'il perde sa principale source de revenus.

des plateformes d'intermédiation, qui se chargent simplement de mettre en relation un fournisseur de services avec un client. Ce n'est pas le sujet ! Sont bien visées les plateformes numériques de travail, qui font appel à des travailleurs

fait mine de se réinventer en leur imposant un statut de tâcheron, comme il y a deux siècles ». Un travailleur indépendant est libre de choisir la façon dont il mène son activité. Il exerce à son compte une activité économique et en supporte les risques. Ce n'est pas le cas des travailleurs des plateformes numériques dont nous parlons, qui sont constamment contrôlés par les algorithmes. Il ne s'agit donc pas de travail indépendant, puisque la dépendance économique et la subordination sont à présent attestées.

Les plateformes doivent respecter les règles du jeu, à l'image des entreprises traditionnelles, mais il n'est pas question de choisir entre salariat et travail indépendant,

Nous souhaitons au contraire ouvrir un débat sur le renforcement de ces deux statuts : le travail indépendant, auquel nous voulons accorder davantage de protection, et le salariat, qui devrait acquérir une plus grande autonomie pour sortir des situations d'asservissement résultant de pratiques managériales abusives. Plus largement, ce texte constitue un jalon important dans le débat sur l'avenir du travail sous toutes ses formes. En effet, l'économie numérique va ouvrir la voie à de nouvelles formes de travail qui se répercuteront sur des pans entiers de la société. Nous avons la possibilité d'influer sur la direction à prendre. Souhaitons-nous tirer vers le bas l'ensemble des statuts professionnels et aboutir à une plus grande précarisation du travail ? Voulons-nous, au contraire, nous engager de façon forte pour que chaque personne puisse s'accomplir librement et en sécurité dans son activité professionnelle ? Nous vous proposons de prendre la voie la plus juste, qui est aussi la plus attendue par les premiers concernés, car le progrès technologique doit avant tout servir les êtres humains, et non les asservir. La

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi de Pascal Savoldelli, que j'ai cosignée avec les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, vise à créer un statut protecteur de certains travailleurs, qui, depuis l'apparition des plateformes numériques, restent des oubliés du droit du travail et de la protection sociale.

Issue du constat que les plateformes de travail sont non pas de simples intermédiaires, mais des organisations productives s'inspirant, plus encore que les entreprises traditionnelles, des logiques de concurrence qui gouvernent le marché, cette proposition de loi tend à adapter le droit du travail à cette situation, afin d'intégrer ces travailleurs dans le salariat. Si la commission des affaires sociales n'a pas adopté ce texte, ce que je regrette, elle a une nouvelle fois reconnu la nécessité d'améliorer les protections dont peuvent bénéficier ces travailleurs. Il convient tout d'abord de rappeler ce qui fonde la distinction traditionnelle entre le salariat et le travail indépendant. La relation entre celui qui possède les moyens de production et celui qui loue sa force de travail est par nature déséquilibrée. Le salarié est en effet placé dans une relation de subordination vis-à-vis de son employeur, dont il dépend pour ses moyens de subsistance. Afin de remédier à ce déséquilibre, le droit du travail a progressivement construit un socle de garanties protégeant les salariés, notamment en matière de rémunération, de temps de travail et de droit au repos. Par ailleurs, le préambule de la Constitution de 1946 garantit aux travailleurs certains droits sociaux et permet ainsi la défense collective de leurs intérêts.

Le droit à une couverture santé complémentaire est également garanti à tous les salariés depuis 2016. Enfin, les salariés sont affiliés de droit à l'assurance chômage, qui leur offre une protection contre le risque de perte de leur emploi. leur emploi. Les protections offertes par le statut de salarié sont principalement garanties et financées par les employeurs ; d'autres constituent des limitations à leur pouvoir de direction. Dès lors, les stratégies consistant à assimiler une relation de travail à une prestation de services fournie par un travailleur indépendant sont aussi anciennes que le droit du travail. Face à ces tentatives, la jurisprudence affirme clairement que la nature de la relation de travail est d'ordre public et ne dépend pas de la qualification qu'en font les parties. Pour apprécier l'existence d'un lien de subordination, le juge se base sur un faisceau d'indices : d'une part, l'autorité et le contrôle exercés par le donneur d'ordre et, d'autre part, les conditions matérielles d'exercice de l'activité. Par exemple, le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé peut constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination. Si celui-ci est démontré, le juge peut requalifier en contrat de travail ce qui était présenté comme un contrat de prestation de services. Les possibilités offertes par le numérique ont donné une nouvelle actualité à ce problème ancien. Si chacun pense aux chauffeurs de VTC et aux livreurs à deux-roues, les plateformes sont présentes dans un nombre croissant de secteurs. Ainsi, elles interviennent dans le placement de travailleurs temporaires, contournant les règles imposées au secteur de l'intérim. Force est de constater que, en réalité, ces plateformes jouent souvent un rôle essentiel dans l'organisation des prestations qu'elles proposent. Ainsi, dans le domaine de la mobilité, les travailleurs ne sont généralement pas en mesure de fixer le prix de la prestation qui leur est proposée. Le tarif est déterminé par un algorithme dont ils ignorent les paramètres. En outre, ils ne connaissent pas toujours à l'avance la destination de la course qu'on leur demande de réaliser et sont tenus de respecter des règles imposées par la plateforme. Enfin, alors qu'en principe un indépendant n'est pas juridiquement subordonné à son client, le non-respect par ces travailleurs des directives données par les plateformes les expose à des sanctions pouvant aller jusqu'à la déconnexion, c'est-à-dire à une forme de licenciement arbitraire. En somme, ces travailleurs connaissent tous les inconvénients de l'indépendance sans en avoir les avantages. Dès lors, des juges ont été amenés à requalifier en contrat de travail la relation entre des travailleurs et des plateformes numériques. Au vu des récents arrêts rendus par la Cour de cassation, on ne peut contester qu'une tendance à l'assimilation au salariat du statut de ces travailleurs se dessine. Toutefois, laisser les juges requalifier au cas par cas des situations individuelles ne saurait constituer une réponse satisfaisante au regard des dégâts causés par ce modèle. Les travailleurs de plateformes portent en germe une nouvelle classe de travailleurs précaires. Certes, ils sont encore peu nombreux- entre 100 000 et 200 000 personnes, selon les estimations -, mais leur nombre a tendance à croître à mesure que se développe l'« ubérisation » de notre société. Surtout, comme le rappelle la crise sanitaire que notre pays traverse, les travailleurs des plateformes font partie des employés les plus exposés de notre économie. Les revenus qu'ils perçoivent, notamment les livreurs à vélo, sont souvent dérisoires. Si le chiffre d'affaires affiché par les chauffeurs VTC est plus important, il ne leur permet pas toujours de couvrir leurs charges. En plus d'être faiblement rémunérés, les travailleurs de plateformes sont nombreux à ne bénéficier ni d'une assurance contre les accidents du travail, pourtant fréquents chez les usagers de la route, ni d'une complémentaire santé. Ce phénomène est la suite logique d'une recherche continue de flexibilité, ainsi que du mouvement général d'externalisation, qui fait sortir de l'entreprise les travaux jugés non rentables jusqu'à transformer les salariés en entrepreneurs faussement indépendants. Il pourrait donc non seulement connaître un développement exponentiel dans certains secteurs, mais encore s'étendre à de nouveaux domaines jusqu'ici épargnés, comme le montre le projet de certains groupes bancaires d'expérimenter l'emploi de conseillers indépendants. Cette évolution a pour corollaire de faire peser toujours davantage le risque économique sur les travailleurs. Face à cette tendance, on assiste cependant à l'émergence d'îlots de résistance. Malgré leur éloignement spontané du syndicalisme et une certaine culture de l'immédiateté, ces travailleurs sont susceptibles de se mobiliser, à l'image du mouvement concerté des livreurs Deliveroo, en juillet 2019, face à la modification de la politique tarifaire de la plateforme. Un mouvement de fond émerge : l'organisation croissante de ces travailleurs. Certaines associations, telles que le Collectif des livreurs autonomes parisiens, le CLAP, se sont ainsi constituées depuis plusieurs années ; elles ont acquis une forme de reconnaissance de la part des plateformes. Par ailleurs, plusieurs organisations syndicales de salariés ont entrepris de s'intéresser aux travailleurs de plateformes. Enfin, des tentatives de structuration des collectifs existants se dessinent. Il n'en reste pas moins que ces tentatives se heurtent à l'absence de reconnaissance législative d'une représentation des travailleurs de plateformes, ainsi qu'au manque de règles structurant le dialogue social. À cet égard, les instances de concertation mises en place par certaines plateformes ne doivent pas faire illusion. Par ailleurs, des initiatives se développent sur le terrain pour proposer un modèle alternatif à celui que promeuvent les grandes plateformes. Elles prennent notamment la forme de sociétés coopératives fondées sur une gouvernance démocratique et un partage équitable des résultats. Face à cette situation, le législateur a jusqu'à présent réagi de manière timide. Le principe d'une responsabilité sociale des plateformes, institué par la loi Travail du 8 août 2016, se traduit par la prise en charge par les plateformes des cotisations d'assurance volontaire contre le risque d'accident du travail, de la cotisation à la formation professionnelle et des frais liés à la validation des acquis de l'expérience. Cette loi a par ailleurs créé un embryon de droit syndical et de droit de grève au bénéfice de ces travailleurs. La loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 est allée dans le même sens, en donnant notamment aux plateformes de mobilité la possibilité d'élaborer des chartes déterminant les conditions et les modalités d'exercice de leur responsabilité sociale. Ces avancées témoignent d'une certaine prise en compte de la situation des travailleurs concernés. Toutefois, elles demeurent largement tributaires du bon vouloir des plateformes elles-mêmes. Surtout, elles tendent à consacrer le recours à des travailleurs indépendants pour des tâches qui pourraient être réalisées par des salariés. de loi crée donc une nouvelle forme de contrat de travail applicable aux travailleurs de certaines plateformes numériques, à savoir celles pour lesquelles la mise en relation est non pas l'objet de l'activité, mais la modalité d'accès et de réalisation du service. Il s'agit notamment, de mon point de vue, des principales plateformes du secteur des transports. Les dispositions du code du travail seraient largement applicables à ces travailleurs, sous réserve de certains aménagements. Le texte laisse une large place à la négociation collective. Ainsi, les modalités de construction et de gestion des emplois du temps et les modes de calcul de la rémunération feraient l'objet d'une négociation annuelle avec les représentants des travailleurs. L'article 2 prévoit l'affiliation obligatoire des travailleurs de plateformes au régime général de la sécurité sociale. En outre, il étend à ces travailleurs le bénéfice de l'assurance chômage. à l'article 4, il complète les dispositions du code du travail applicables aux travailleurs indépendants des plateformes. Il élargit ainsi la possibilité d'assurance des travailleurs à la charge de la plateforme, en mentionnant les maladies professionnelles, et tend à laisser aux travailleurs le choix d'adhérer ou non au contrat collectif proposé par la plateforme. L'objet de cette proposition de loi est donc bien de trancher clairement, dans la lignée des récents arrêts de la Cour de cassation, en faveur d'une assimilation à des salariés de ces travailleurs considérés comme des indépendants alors qu'ils n'ont pas la pleine maîtrise de leur travail, ce dont quelques grandes entreprises

mesdames, messieurs les sénateurs, je veux avant tout remercier le groupe communiste républicain citoyen et écologiste d'avoir fait inscrire à l'ordre du jour du Sénat la proposition de loi de M. Savoldelli, car il a mené un travail très important et empreint de l'engagement fort que nous lui connaissons. connaissons. Nous partageons tous, me semble-t-il, un même constat : l'essor de l'économie des plateformes numériques de mise en relation des travailleurs avec les consommateurs est l'une des évolutions les plus importantes du marché du travail depuis une dizaine d'années. D'ailleurs, dans le cadre du confinement, cette évolution s'est révélée constituer un maillon à la fois important et fragile. Aussi, la double crise, sanitaire et économique, que nous traversons pose avec une acuité renforcée la question des protections sociales et économiques dont ont besoin ces acteurs particulièrement exposés.

En effet, appréhender l'impact pluridimensionnel- économique, social et territorial -de cette évolution mondiale est d'autant plus complexe qu'il existe- vous le savez, vous l'avez partiellement rappelé -une grande variété de structures et une multiplicité d'acteurs aux aspirations très diverses. Cela a d'ailleurs été parfaitement souligné lors de l'examen de ce texte par votre commission des affaires sociales, mais aussi dans le rapport de la mission d'information conduite par Mmes Catherine Fournier et Frédérique Puissat et M. Michel Forissier, rapporteur de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, que je salue à cette occasion.

En d'autres termes, le développement pérenne de ces activités ne doit pas être synonyme de trappe à précarité ou de dumping social, mais doit constituer un vrai tremplin vers un emploi de qualité ; il doit être doté de garanties sociales solides et nouvelles. Depuis 2016, le législateur s'efforce de construire la responsabilité sociale des plateformes en la ciblant sur celles d'entre elles qui fixent les prix et déterminent les conditions d'exécution des prestations.

permet de renforcer le droit à la formation professionnelle des travailleurs des plateformes en définissant notamment des règles d'alimentation renforcée du compte personnel de formation. Je rappelle par ailleurs que cette loi a mis en place un socle d'obligations, le droit à la déconnexion et la transparence quant au prix des courses pour les plateformes électroniques de mise en relation avec des chauffeurs de VTC et des coursiers. S'agissant des chartes homologuées par le ministère du travail, elles ont vocation à inciter les plateformes à être plus transparentes quant à leurs engagements sociaux, tout en leur laissant la possibilité d'aller plus loin. Enfin, concernant le volet du dialogue social, les débats parlementaires ont fait clairement émerger la nécessité d'organiser une meilleure représentation des travailleurs ; je partage C'est un point déterminant : au-delà du socle des droits garantis par les dispositifs législatifs, l'émergence de droits nouveaux correspondant aux réelles aspirations de ces travailleurs ne pourra résulter que de l'organisation d'un dialogue social équilibré et durable. Cela suppose un nouveau modèle de représentation de ces travailleurs. C'est précisément l'objet de l'ordonnance prévue à l'article 48 de la loi d'orientation des mobilités. Dans la perspective de son élaboration, le Gouvernement a confié en janvier dernier une mission à M. Jean-Yves Frouin, ancien président de la chambre sociale de la Cour de cassation, appuyé par un groupe d'experts. de loi aborde l'ensemble des questions pertinentes au sujet de ces nouvelles formes d'emploi, tous les défis que nous devons relever pour favoriser une économie des plateformes à la fois créatrice d'emplois et socialement responsable

Nous sommes conscients que le cadre législatif actuel ne permet pas de répondre pleinement à l'ensemble de ces défis. Il faut donc aller plus loin et construire une réponse adaptée à chacun de ces enjeux. Malheureusement, il n'y a pas de solution unique, facile et uniforme qui réponde à l'ensemble des enjeux ; si une telle solution existait, gageons qu'elle aurait déjà été adoptée par l'ensemble des États, tous confrontés aux mêmes mutations.

Il lui appartiendra dans les tout prochains mois de formuler des propositions sur chacune des problématiques posées par cette nouvelle forme d'emploi ; il pourra s'appuyer sur les débats de ce matin, et nous lui demanderons Le fruit de ses travaux devra nous aider à construire ensemble un chemin certes étroit, mais possible pour renforcer de manière pérenne le socle des droits dont doivent bénéficier les travailleurs des plateformes, sans remettre fondamentalement en cause la souplesse apportée par le statut d'indépendant.

Je les invite d'ailleurs, s'ils le souhaitent, à continuer de contribuer aux travaux que nous mènerons sur ce sujet dans les prochains mois. Enfin, parce que cette problématique dépasse le simple cadre national, nous continuons à la pousser à l'échelon européen. c'est sous l'impulsion de la France que la Commission européenne s'est engagée à préparer une initiative européenne pour établir des conditions de travail justes pour les travailleurs des plateformes et améliorer leur accès à la protection sociale.

à laquelle nous sommes, en tant que parlementaires, spécialement sensibles. Ces dernières années, de nouvelles formes de travail se sont développées avec l'essor des nouvelles technologies de l'information, qui permettent la mise en relation de millions d'utilisateurs en temps réel. Les plateformes numériques ont en commun de servir d'intermédiaires entre travailleurs et clients, équilibrant l'offre et la demande au moyen d'algorithmes et ouvrant le champ de l'économie collaborative à l'échelle mondiale.

des actifs, ces travailleurs sont en forte croissance dans de multiples secteurs, comme l'hôtellerie, les transports, la banque ou le secteur juridique. Les plateformes concurrencent l'offre traditionnelle de services, encadrée par un droit du travail plus protecteur, et offrent de nouvelles perspectives d'emploi à des personnes éloignées du marché du travail, essentiellement des jeunes, dans un contexte de chômage élevé. Des difficultés d'interprétation juridique se posent lorsque ces travailleurs indépendants sont économiquement dépendants. au-delà de la simple fonction d'interface, certaines plateformes organisent le temps de travail, la rémunération et les conditions de mises en relation, hiérarchisant les contenus selon les utilisateurs. Le niveau d'intervention de ces plateformes et l'importance des revenus tirés de leur activité justifient l'attention que nous leur portons.

La réflexion que nous menons actuellement devrait bénéficier à l'ensemble des indépendants, dont le régime de protection sociale n'est pas aussi complet que celui qui s'applique dans le cadre du salariat- pour avoir été longtemps avocat, je sais de quoi je parle ... Les

Je ne pense pas qu'il soit pertinent d'ajouter un nouveau niveau de complexité administrative, source d'insécurité juridique. En revanche, il paraît opportun d'offrir à ces travailleurs l'accès à une complémentaire santé et à une couverture des accidents du travail et maladies professionnelles, en particulier pour les plus exposés à ces risques.

Il importe également de poser les conditions d'un dialogue entre les plateformes et les travailleurs autour des algorithmes utilisés, lorsqu'ils déterminent de façon importante les conditions de travail et de rémunération. Il s'agit de trouver un juste équilibre entre la liberté d'entreprendre et le besoin de protection, étant entendu qu'un statut trop rigide risquerait de limiter les opportunités d'emploi offertes à de nombreux travailleurs. Faut-il aller vers une segmentation plus marquée du droit du travail ou, au contraire, une convergence des droits entre travailleurs salariés et indépendants au sein d'un droit de l'activité professionnelle ? La question reste ouverte.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, depuis quelques années, les centres urbains ont vu émerger une nouvelle catégorie de travailleurs, spécialisés dans le service aux habitants recherchant une offre de transport ou de livraison personnalisée à coût très compétitif. La vision de ces coursiers à vélo ou en voiture alerte sur ce nouveau modèle d'organisation du travail : dans quelles conditions ces intervenants exécutent-ils leurs missions, comment sont-ils dirigés et sur quels critères repose leur rémunération ? ? Mes collègues Michel Forissier, Frédérique Puissat et moi-même nous sommes intéressés à ce dossier de manière plus générale : nous avons été chargés par la commission des affaires sociales d'une mission d'information sur le droit applicable aux travailleurs indépendants économiquement dépendants. Après six mois de travaux et plus de quarante auditions, nous avons rendu notre rapport la semaine dernière, certains que les plateformes numériques ne se résument pas à celles des livreurs et des coursiers. des coursiers. Nous y rappelons que l'apparition des plateformes numériques de mise en relation a donné une acuité nouvelle à la question, relativement classique, de la frontière entre salariat et travail indépendant. Instaurer une présomption de non-salariat pour l'ensemble des travailleurs utilisant une plateforme conduirait à valider des stratégies de contournement du droit du travail, au détriment des travailleurs. À l'inverse, qualifier de salariés, par voie législative, des travailleurs qui demeurent libres d'organiser leur travail sans être soumis à un pouvoir de direction de la part de la plateforme poserait un certain nombre de problèmes juridiques. Au demeurant, le salariat n'apparaît pas comme une revendication majoritairement partagée par les travailleurs concernés. Nous touchons là à un modèle de société décloisonnée réclamé par les nouvelles générations, qui y trouvent plus d'indépendance et de liberté. À charge pour nous d'étudier les moyens de protection sociale associés. En particulier, nous devons dépasser la question du statut et universaliser certains droits sociaux. Mes collègues rapporteurs de la mission d'information et moi-même avons distingué quatre types de plateformes. Premièrement, des plateformes de services organisés fournissent des prestations hors ligne standardisées, délivrées par des professionnels, notamment dans les secteurs de la conduite- Uber, Kapten, Bolt -et de la livraison de marchandises- Deliveroo, Uber Eats, Stuart. Deuxièmement, des plateformes de placement ont pour objet la mise à disposition de travailleurs indépendants auprès d'entreprises pour des missions ponctuelles. Ces intermédiaires peuvent déterminer le prix des prestations, mais n'interviennent pas ou peu pour organiser les tâches, qui sont définies en amont. Troisièmement, les plateformes dites de mise en relation entre des travailleurs indépendants et des clients sont des plateformes de, comme Malt, qui présentent des travailleurs indépendants qualifiés à des entreprises. la plateforme ne fixe pas le prix et n'interfère pas dans la négociation ; elle touche une commission évaluée sur la prestation fournie. Quatrièmement, les plateformes de microtravail renvoient au développement de l'externalisation l'externalisation de tâches fortement fragmentées et à faible valeur ajoutée ; il s'agit notamment d'Amazon Mechanical Turk.

Ce nouveau modèle d'entreprise s'organise, se développe et contrôle ses échanges grâce à un seul outil : l'algorithme. Celui-ci, qu'on pourrait appeler le bras armé des plateformes, protégé, car relevant du secret industriel,

de pouvoir agir sur l'algorithme, il nous reste à oeuvrer sur les conditions de travail et la couverture sociale des travailleurs qui en dépendent. L'écho médiatique laisse entendre que cette nouvelle organisation du travail

Jusqu'à présent, le législateur n'a pas tranché : il a laissé les juges utiliser les outils disponibles et appliquer la conception classique du droit travail en vigueur, reposant sur le lien de subordination constitutif d'une relation salariée.

l'article 1 transforme la relation commerciale du travailleur indépendant de plateforme en un contrat relevant du droit du travail. Cette hypothèse, centrée sur les plateformes de services, est trop restrictive et fait fi de la diversité des plateformes numériques.

vous avez annoncé, le 5 mars dernier, le lancement d'une mission sur le statut des travailleurs de plateformes numériques. Au nom de mes collègues, je souhaite vivement que l'ensemble des débats et travaux parlementaires nourrissent cette vaste réflexion, comme vous venez de nous le proposer. La parole est à M. Michel Forissier.

Nous pouvons être collectivement fiers que le Sénat travaille, depuis maintenant deux ans, sur la situation des travailleurs indépendants des plateformes numériques, car le débat est à la fois social et économique la protection des travailleurs de ce nouveau modèle économique mondial est une question d'accompagnement de la mutation socioéconomique pour éviter le piège de la précarité. Je remercie Mme la rapporteure de soutenir ce matin cette discussion si importante, afin que nous partagions nos réflexions. La diversité des situations des travailleurs indépendants des plateformes numériques implique que le législateur réfléchisse au-delà de la simple requalification en contrat de travail. Les travailleurs des plateformes exercent un travail indépendant, défini en opposition au salariat classique,

Les travailleurs des plateformes sont visibles partout, sauf dans les statistiques : il n'existe guère de recensement exhaustif, mais les chiffres des travaux menés vont de 100 000 à 200 000 personnes.

Les travaux de l'Insee indiquent que 4 % de l'ensemble des indépendants sont économiquement dépendants d'un intermédiaire, qui n'est pas nécessairement une plateforme. Les profils des travailleurs des plateformes sont hétérogènes, allant de l'étudiant à vélo qui transporte des repas au chauffeur de VTC qui exerce cette activité à titre principal, en passant par le travailleur qualifié bien rémunéré et parfaitement autonome qui recourt à des plateformes pour trouver ses clients. Les plateformes numériques sont elles-mêmes des structures diverses- certaines sont des multinationales ; je vous fais grâce des détails, car vous les connaissez. Proposer à ces travailleurs un statut à mi-chemin entre le salariat et le régime indépendant tout en introduisant de nouveaux droits sociaux n'est pas souhaitable

Par hypothèse, les travailleurs indépendants des plateformes numériques bénéficient de la même couverture sociale que les ressortissants du régime général pour ce qui est de la santé et des prestations de la branche famille, décorrélées du statut. Toutefois, les indépendants ne relèvent pas du droit du travail et ne bénéficient pas

Les travailleurs indépendants des plateformes numériques sont souvent désarmés face aux accidents et à la rupture de la relation de travail. La période que nous traversons, avec l'épidémie et ses conséquences sanitaires et économiques, rend plus que jamais visible le besoin de protection de certains d'entre eux, parfois dans des situations très

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la question du statut des travailleurs de plateformes numériques est malheureusement destinée à nous occuper longtemps ; elle est symptomatique d'une forme de capitulation à tous les niveaux, y compris à Une réalité sociale et économique se déploie : elle correspond à un modèle alternatif à celui qui fonde notre pacte social. Ce nouveau modèle est très « ancien monde », puisqu'il obéit à des logiques d'asservissement par la misère et l'exploitation. Il s'impose de nouveau, sans être pour autant ni explicité ni soumis à validation démocratique. Le sort fait aux travailleurs des plateformes numériques est une manifestation de ce glissement, qui menace de virer en dégringolade. Le clinquant de technologies sophistiquées sert- difficilement -de voile à la réinstallation de logiques passéistes, que les luttes sociales nous avaient permis de dépasser. Nous renouons avec le tâcheronnage Malheureusement, ici comme ailleurs, les systèmes destructeurs reprennent force et repartent à l'offensive à la moindre faiblesse comme à la moindre négligence ... Nadine Grelet-Certenais, Olivier Jacquin et moi-même avons défendu dans cet hémicycle une proposition de loi visant à rétablir les droits sociaux des travailleurs numériques. Affinée en séance, elle avait pour objet de rappeler les vertus aujourd'hui indépassées du salariat. Il s'agissait d'en imposer le recours au profit de travailleurs victimes de donneurs d'ordre qui tirent profit des angles morts de notre législation et d'un rapport de force extraordinairement déséquilibré. Nous avions promu les solutions prévues par le code du travail, en réhabilitant le contrat de travail et en soutenant le recours aux coopératives d'activité et d'emploi. En particulier, la valorisation du coopérativisme, un mouvement dont il faut soutenir le développement dans le cadre d'une indispensable économie sociale et solidaire, est un enjeu clé.

il lui faut un cadre protecteur, d'autant plus que les travailleurs de plateformes sont membres d'une profession habituée à un très fort turnover, ce qui est une difficulté supplémentaire.

ne va pas suffisamment à la reconquête du terrain perdu pour les droits des travailleurs, au moment même où, en France et dans le reste du monde, les décisions de justice touchant aux travailleurs de plateformes tendent à réhabiliter le salariat.

on laisserait aux personnes le soin de concéder ou d'obtenir d'hypothétiques avancées sociales, sans que la puissance publique puisse suffisamment jouer son rôle de garante. En fait, j'ai l'impression que ce que nous essayons tous de proposer relève d'une forme d'impuissance devant un phénomène massif et qui s'étend aujourd'hui à de nombreux secteurs. Pourtant, le droit du travail n'a pas à se soumettre aux logiques économiques : il doit au contraire s'imposer à elles et les façonner

Mes chers collègues, la présente proposition de loi et l'ensemble des débats sur les travailleurs de plateformes montrent singulièrement que nous devons repenser la place de la valeur travail dans notre société : le travail doit servir les travailleurs et permettre leur émancipation, une émancipation dont nous sommes actuellement très loin

ce genre existent principalement dans les domaines du transport de personnes, de la livraison de repas ou de marchandises, des services à la personne et de petits emplois : la seule limite est la créativité des concepteurs concepteurs ... S'agissant des rapports entre les travailleurs et les plateformes, le droit a aussi son mot à dire. Deux décisions de la chambre sociale de la Cour de cassation, du 28 décembre 2018 et du 4 mars 2020,

soulevant de nombreuses interrogations, y compris de votre part, madame la ministre : dès le lendemain, vous avez annoncé la création d'une mission conjointe avec le ministre de l'économie et des finances sur les travailleurs des plateformes numériques, leurs droits et leurs protections. Certains manques ont servi de base à la chambre sociale de la Cour de cassation dans les deux arrêts que je viens de citer. Ainsi, du fait de leur statut d'autoentrepreneur, les travailleurs des plateformes numériques ne bénéficient d'aucune protection sociale ; en cas d'accident du travail, pas de protection digne. Les assurances proposées par les plateformes sont souvent insuffisantes, quand elles ne sont pas complètement inopérantes : l'une n'assure pas le torse des livreurs à vélo, l'autre pas les viscères d'un livreur qui, accidenté lors d'une livraison, a vu son abdomen perforé ... Voilà pourquoi il est urgent de travailler sur cette question et d'offrir à ces travailleurs de vraies protections. La technologie a évolué plus vite que notre droit. Il existe une zone de vide juridique entre le statut de salarié et le statut d'indépendant.

Si l'objectif est louable, il convient néanmoins de s'interroger sur la pertinence de créer une nouvelle forme de contrat de travail applicable aux travailleurs de certaines plateformes numériques. Ces travailleurs forment un public disparate : certains indépendants sont tout à fait à l'aise avec les conditions d'exercice imposées par les plateformes et s'adaptent à ce modèle. Ceux-là n'aspirent pas nécessairement à être dotés d'un statut qu'ils pourraient juger trop strict au regard de la flexibilité que leur offre leur qualité d'indépendants. D'autres-les plus précaires-, ceux qui exercent cette activité afin d'en tirer un complément de revenus ou sur des périodes plus courtes, souhaiteraient davantage de protection sociale,

consensus. Des convergences existent par ailleurs- et c'est heureux -sur la nécessité de mettre en place un filet de sécurité commun qui s'adresserait tant aux plus précaires qu'aux indépendants pouvant connaître des accidents de parcours.

qui permettent d'améliorer les protections des travailleurs et leurs relations avec les plateformes, notamment en matière de dialogue social. Il faut agir vite, car le futur s'écrit déjà. Quand la voiture autonome sera mise au point, lorsque nos livraisons de repas et de biens pourront se faire de manière automatisée, que deviendront les femmes et les hommes qui aujourd'hui sont chargés de nous transporter et de livrer nos commandes ? Quelles garanties de formation, de reclassement, d'évolution professionnelle ou de réorientation pourront leur être proposées ? Comment accompagner ces travailleurs, pour les sortir de ces « trappes à précarité », et leur permettre de ne pas dépendre uniquement d'un modèle économique qui, à terme, se retournera contre eux ?

Pour autant, ce texte est une contribution importante, et j'espère que le Gouvernement saura entendre certains arguments qui sont présentés. La parole

La crise sanitaire de la Covid-19 n'a fait que renforcer la nécessité pour la commission des affaires sociales de se pencher sur la situation de ces travailleurs bien souvent désarmés face aux accidents et au fonctionnement des algorithmes des plateformes. Les derniers travaux en date sont le fruit de la réflexion d'une mission d'information relative au droit social applicable aux travailleurs indépendants économiquement dépendants, qui a rendu officiellement ses conclusions le 20 mai. Le rapport rédigé par mes collègues Forissier, Fournier et Puissat liste une série de quatorze recommandations pour améliorer la situation des travailleurs des plateformes économiques, prenant ainsi en compte la diversité des situations. La plupart des recommandations consistent à étendre, dans la droite ligne des précédentes lois en la matière, notamment la loi d'orientation des mobilités, le bénéfice des garanties qu'offre le code du travail. Au total, entre 100 000 et 200 000 personnes seraient concernées. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour examiner un texte déposé par le groupe CRCE au mois de septembre. Nous ne saurions débattre d'une proposition de loi relative aux droits sociaux des travailleurs numériques sans rappeler le contexte dans lequel ces derniers évoluent. Les travailleurs des plateformes représentent environ 0,8 % de la population active. Ils se répartissent entre trois catégories de travailleurs : les travailleurs, par ailleurs salariés, qui utilisent les plateformes afin de compléter leurs revenus les travailleurs indépendants qui recourent aux plateformes comme forme d'activité exclusive- le rapport d'information fait état de travaux de l'Insee selon lesquelles 4 % des indépendants, soit 0,5 % de la population active occupée, sont économiquement dépendants d'un intermédiaire, qu'il s'agisse ou non d'une plateforme enfin, les travailleurs indépendants hautement qualifiés qui souhaitent bénéficier de davantage de flexibilité en se tournant vers un intermédiaire numérique, comme les, dont le principal atout est la simplification des démarches administratives. Les récentes lois ont permis d'instituer une responsabilité sociale des plateformes au bénéfice des travailleurs indépendants, mais également d'approfondir cette démarche de régulation de la relation entre les plateformes numériques et les travailleurs indépendants- je pense à la prise en charge, plafonnée par décret, de la cotisation du travailleur pour une assurance couvrant le risque d'accident du travail, au droit d'accès à la formation professionnelle continue et au bénéfice de la validation des acquis de l'expérience, aux droits collectifs tels que la protection des travailleurs participant à des mouvements en vue de la défense de leurs revendications professionnelles, ou encore à la faculté, pour les travailleurs visés, de constituer une organisation syndicale. Ces avancées ne sont qu'un début dans la régulation des relations avec les plateformes numériques, dont la nouveauté met en question les catégories juridiques existantes et implique une réflexion approfondie. Cet encadrement des relations est actuellement renforcé, mais nous devons garder à l'esprit l'objectif de concilier l'indépendance de ces travailleurs, le modèle économique des plateformes et la protection des droits sociaux.

Ce statut intermédiaire n'est pas souhaitable, car il entraînerait des effets contraires aux objectifs visés. Pour autant, cette proposition de loi soulève des éléments très importants : la représentation des travailleurs numériques et les algorithmes. Cela peut paraître un peu abstrait pour certains d'entre nous, mais l'objectif des plateformes est de constituer un intermédiaire dont le rôle est de créer de la valeur en facilitant des transactions au moyen d'algorithmes de recherche, d'appariement, de paiement, etc., qui lui sont propres. Si les algorithmes ont un rôle déterminant dans le fonctionnement des plateformes, ils rendent également celles-ci plus opaques. Ils peuvent, par exemple, entraîner certaines discriminations, tarifaires entre autres, que nous devons prendre en compte, afin que les travailleurs du numérique puissent disposer de toutes les clés de compréhension et travailler en toute connaissance de cause avec ces intermédiaires que constituent les plateformes. C'est pourquoi le Premier ministre a confié, le 14 janvier dernier, à Jean-Yves Frouin, ancien président de la chambre sociale de la Cour de cassation, une mission visant à définir les différents scénarios envisageables pour construire un cadre permettant la représentation des travailleurs des plateformes numériques. Cette mission est chargée de préparer l'ordonnance prévue par l'article 48 de la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019, qui doit déterminer les modalités de la représentation de ces 200 000 travailleurs de plateformes. Comme vous venez de l'annoncer, madame la ministre, le périmètre de cette mission sera élargi. la question non seulement de la représentation des travailleurs du numérique, mais aussi de la transparence des modes de fonctionnement des plateformes, autrement dit les algorithmes, et d'autres compétences économiques, numériques et juridiques. L'objectif reste inchangé : renforcer le droit de ces 200 000 Français. Il est donc indispensable d'en attendre les résultats. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, les réponses présentées dans cette proposition de loi ouvrent des pistes. Nous en remercions les auteurs, mais ces pistes ne répondent pas aux vastes problèmes posés par le développement de l'économie des plateformes numériques. Pour cette raison, le groupe La République En Marche votera contre ce texte.

Je remercie enfin mes collègues Fournier, Puissat et Forissier de la qualité de leur rapport. Même si nous ne partageons pas les préconisations formulées, le rapport dresse un état des lieux largement partagé. en cause se répand à tous les secteurs de la société, souvent au détriment des travailleuses et travailleurs les plus précaires, comme les aides ménagères, mais aussi des entreprises vertueuses. Au cours du travail d'élaboration du texte, avons été bousculés par nos rencontres avec les livreuses et les livreurs, car il s'agissait parfois de jeunes hostiles au salariat, dégoûtés par leur expérience et par celle de leurs parents, maltraités par un management avilissant, et, en conséquence, à la recherche d'une grande autonomie de travail et d'une sortie de la précarité. Au départ, ils ont été séduits, parfois, par la liberté vantée par les plateformes. Mais où est la liberté lorsqu'on travaille sept jours sur sept et dix heures par jour pour moins que le SMIC horaire ? En détournant le statut d'autoentrepreneur en salariat déguisé pour échapper à leurs obligations en termes de salaire et de protection sociale, Uber, Deliveroo et toutes ces grandes plateformes ne proposent en réalité la liberté d'exploiter. Les maîtres de forges ont été remplacés par un iPhone avec une application et des algorithmes, mais la réalité est la même : ce sont les nouveaux forçats du travail. Si Victor Hugo devait réécrire aujourd'hui, assurément Cosette livrerait des repas à vélo, les Thénardier seraient l'une de ces grandes multinationales, et je ne sais pas encore qui tiendrait le rôle de Javert, madame la ministre, tant nous tardons à légiférer pour faire respecter le droit du travail. C'est pourquoi

et, d'autre part, en permettant de rendre efficiente une véritable autonomie, existante en droit du travail, mais qui s'est délitée. L'objectif n'est pas d'accompagner ou d'adapter l'ubérisation de la société, ni de créer pour les travailleurs des plateformes un troisième statut d'indépendants économiquement dépendants. Les plateformes visées sont les plateformes de travail, celles qui font semblant d'être des plateformes de mise en relation entre des indépendants et des clients, mais qui, en réalité, font tout autre chose elles adoptent cette posture d'intermédiaire pour nier l'exercice sur les travailleurs d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction qui supposerait l'application de la législation sociale.

ont donc pris des risques pour leur santé en travaillant sans matériel de protection, et ils ont été obligés d'improviser eux-mêmes des règles. Or ces plateformes ne sont pas neutres dans la prestation réalisée. Au contraire, comme en témoigne le récent arrêt Uber rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation, ces plateformes organisent et encadrent l'activité des travailleurs. Les prescriptions des contremaîtres ont simplement été remplacées par celle des algorithmes, traduction informatique des directives patronales. Cela n'est pas acceptable ! Ces travailleurs doivent pouvoir jouir des droits qui sont les leurs. Ils doivent bénéficier du droit du travail et de la protection sociale.

Ce texte a vocation à permettre l'application effective du droit social, la mobilisation des travailleurs, mais aussi à lutter contre la dégradation du salariat en garantissant une réelle écoute, une véritable émancipation collective. Nous ne voulons pas laisser les plateformes galvauder et paupériser l'entrepreneuriat. Nous ne voulons pas que la nouveauté d'accès à un service serve de prétexte à certaines entreprises pour faire de la concurrence déloyale à nos entreprises vertueuses, au détriment des plus précaires. La mutation de l'économie, la dépendance des travailleurs comme des entreprises à ces plateformes dont le modèle économique repose sur le non-respect des règles sociales et fiscales, doit nous conduire à nous interroger, car les entrepreneurs sont aussi

Certains ont fait le choix de passer par des organismes respectueux des entrepreneurs comme des travailleurs. N'oublions pas que la livraison est un service, mais surtout un vrai travail. Elle se fait au prix de la sueur du travailleur.

En attendant l'avènement d'une société égalitaire où chaque individu pourra s'épanouir dans son travail, en continuant d'encourager les coopératives de livreurs, comme à Bordeaux, nous proposons de poser une première pierre à l'édifice en accordant un statut et des droits à celles et ceux qui n'en ont pas.

de loi qui nous est présentée aujourd'hui par les membres du groupe CRCE fait suite à plusieurs travaux sur ce qu'il est coutume d'appeler les « travailleurs des plateformes ». Sans chercher à être exhaustive, j'en citerai quelques-uns qui ont déjà été rappelés par des orateurs précédents : la loi Travail de 2016, qui a créé au sein de la septième partie du code du travail un chapitre

aspects que nous avons pu approfondir avec la rapporteure au cours notamment d'auditions toujours très enrichissantes. Dans son article 1, la présente proposition de loi introduit un nouveau livre dans le code du travail consacré aux travailleurs des plateformes et prévoit qu'au statut d'autoentrepreneur et d'indépendant peu se substituer un CDI ou un CDD dont le temps de travail et la rémunération donneraient lieu à une négociation annuelle. Rappelons, tout d'abord, que la multiplicité des plateformes, même si ce texte en limite la portée, comme l'absence de statistiques ou leur faible épaisseur du fait d'un turnover important, ne permettent pas d'affirmer que cette transformation est

L'article 2 de la présente proposition de loi étend le droit à l'assurance chômage, dont l'intérêt est indéniable, mais sans en préciser le financement et en prenant en compte des périodes d'activité qui peuvent paraître complexes à atteindre.

de demander des explications sur des modifications d'algorithme concernant l'organisation et les conditions de travail, et les aiderait à solliciter le recours à un expert spécialiste en algorithmes dont les frais seraient à la charge de la plateforme.

Par ailleurs, force est de constater que l'identification et le recensement des experts spécialistes relèvent de la gageure. Qui sont-ils ? Combien coûtent-ils ? Ont-ils une connaissance spécifique des algorithmes et du droit du travail ? Pourront-ils suivre les évolutions constantes ? Autant de questions auxquelles nous n'avons pas obtenu de réponse au cours des auditions et qui mettent à mal l'efficience du dispositif proposé.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens à mon tour à remercier mes collègues de nous permettre d'approfondir ce débat sur les conditions de travail et d'emploi des travailleurs

offre la possibilité du statut original d'entrepreneur salarié associé. Celui-ci a été inventé en 2014 pour répondre aux besoins de l'économie collaborative et des plateformes,

existant. Ma collègue et moi-même notons avec satisfaction que notre proposition a fait progresser et évoluer la réflexion de nombreux acteurs, à commencer par nos collègues de la majorité sénatoriale, puisque cette solution fait partie des recommandations de leur rapport paru il y a quelques jours.

restreint à certains modèles de plateformes numériques. Dans son principe, le devoir de vigilance mériterait toutefois d'être élargi à l'ensemble du champ de l'économie, dès lors que les modèles économiques peuvent légitimer la présence de travailleurs indépendants. Avec les dérégulations spécieuses que nous connaissons depuis quelques décennies, un donneur d'ordre qui respecte la loi peut malgré lui créer les situations indécentes que nous dénonçons, particulièrement en utilisant le sous-statut d'autoentrepreneur dénoncé dans le récent rapport précité. L'exemple le plus flagrant de cette déresponsabilisation des donneurs d'ordre était excellemment rapporté par le journal lundi soir. L'article dressait le portrait d'un migrant récemment arrivé qui n'était pas payé depuis deux mois. Le travailleur pensait travailler pour la plateforme Frichti alors qu'il travaillait en fait pour un sous-traitant. Or la plateforme affirme ne connaître ni ce sous-traitant ni ce travailleur. Comment est-ce possible ? Vous le constatez, nous proposons un nouvel angle d'attaque pour lutter contre le cyber-précariat et la dictature de l'algorithme. remercie mes collègues du groupe CRCE de nous offrir l'opportunité de débattre et de chercher des solutions à ce cancer qu'est l'ubérisation du travail. Monique Lubin a indiqué notre position de fond Madame la ministre, le confinement a mis en évidence la détresse de nombreux travailleurs surexploités, indépendants fictifs, exposés aux risques de la route et au Covid-19, et ne disposant pas de droits suffisants lorsque l'activité cesse. J'ai déjà eu l'occasion de demander qu'on leur accorde une protection comme s'ils étaient salariés.

social. Mes chers collègues, profitons de l'occasion de ce débat pour dire non aux chartes et aux bricolages gouvernementaux, pour dire non à l'ubérisation du travail. Je terminerai en citant le fondateur de la CAE québécoise, Eva, qui, avec son bel accent, nous disait dans une récente réunion en téléconférence que « l'économie collaborative qui existe doit être socialisée et solidarisée ».

Le numérique a des effets indéniablement importants sur le monde du travail. La dématérialisation des entreprises de services et l'indépendance accrue des travailleurs se heurtent aux formes de travail traditionnel. Ces deux aspects soulèvent la question de l'évolution de la protection des droits des travailleurs au sein de ce nouveau modèle. Derrière le terme vague « ubérisation » se profile une nouvelle configuration du statut de salarié. Cette forme inédite d'emploi questionne certains acquis de notre droit du travail. La liberté octroyée aux travailleurs des plateformes du numérique est parfois un moyen de contourner les structures de protection salariale. En effet, le travailleur, bien que déclaré autoentrepreneur, reste au service d'une structure numérisée. S'il ne faut pas extrapoler la place des travailleurs numériques dans notre économie, il convient de rappeler que ces derniers représentent 1 % du bassin d'emploi Les travailleurs des plateformes du numérique évoluent dans un cadre légal inapproprié. En effet, le code du travail ne reconnaît que deux statuts de travailleur : salarié et travailleur indépendant. Seuls les salariés bénéficient du régime général de la sécurité sociale et de l'assurance chômage. Dès lors, les travailleurs des plateformes du numérique sont exposés à la précarité et ne sont pas en mesure de renégocier leurs conditions de travail. Pour autant, cette prétendue exploitation d'une intensité digne du siècle dernier est-elle systématique du mode de fonctionnement de ces plateformes ? Doit-on soumettre ces entreprises à un régime spécifique extrêmement rigoureux, quitte à les fragiliser ? Il me semblerait plus convenable de faire preuve de raison : la révolution numérique, bien qu'elle ébranle notre conception actuelle du monde du travail, est aussi le terreau et l'incubateur de multiples projets qui enrichissent notre économie. Soyons clairs : certaines plateformes internationales disposent de moyens financiers suffisants pour absorber de nouvelles contraintes, mais ce n'est pas le cas d'autres structures, notamment les jeunes entreprises innovantes françaises, souvent plus vertueuses. Plus encore, les plateformes du numérique sont une véritable porte d'entrée sur le marché du travail pour les travailleurs peu qualifiés. La mise en place de telles restrictions aura des conséquences négatives sur le nombre d'emplois créés par les plateformes du numérique. C'est pourquoi j'estime que la question complexe des plateformes ne peut être résolue par le biais de cette proposition de loi. Raisonner dans la généralité nous empêche de saisir les particularités propres à chacune des plateformes du numérique. Astreindre sous le même régime toutes ces entreprises revient à condamner les plus fragiles. Je tiens à réaffirmer mon engagement pour la protection du statut des travailleurs, et bien que je considère comme souhaitable d'étendre aux travailleurs des plateformes du numérique certaines garanties du code du travail, la méthode n'est pas la plus adaptée. Je tiens notamment à souligner la nécessité de protéger les travailleurs des plateformes numériques contre les ruptures de contrat abusives, et mettre un point d'honneur à garantir une protection à ces derniers. Celle-ci se devra d'être différenciée selon les secteurs et les entreprises. À cet égard, il est de notre ressort d'améliorer la protection sociale des travailleurs des plateformes numériques. Au vu de la crise économique qui se profile, nous ne pouvons toutefois faire peser sur les entreprises de trop fortes contraintes économiques. C'est pourquoi la proposition de loi doit considérer davantage la possibilité pour les travailleurs de souscrire à une assurance relative aux accidents du travail et maladies professionnelles ou à une complémentaire santé. Cette couverture suffit à assurer les frais médicaux afférents à une maladie ou à un accident lié à l'exercice d'une profession. exerçant une profession libérale, les artisans, les commerçants et les infirmiers y ont eux-mêmes recours dans l'exercice de leur profession. Il serait plus opportun de s'intéresser à la rédaction d'une proposition de loi relative aux règles de la microentreprise, afin de mettre celles-ci à jour au regard des nouvelles problématiques que soulève l'émergence de plateformes numériques. J'insiste sur la possibilité d'inclure, lorsqu'un régime d'autorisation préalable serait pertinent, des critères sociaux dans leurs agréments. J'ai la conviction que cela permettrait de rationaliser les conditions de travail des employés de ces plateformes. Par ailleurs, une réglementation plus souple serait davantage susceptible de s'adapter à la diversité de ces dernières. L'essentiel de notre mission est d'instaurer un dialogue apaisé entre les multiples acteurs des plateformes numériques. C'est pourquoi je considère que la création d'instances de dialogue social, où travailleurs indépendants et représentants des plateformes pourraient se rencontrer régulièrement et échanger autour de thèmes prédéfinis,

ce que faisait la puissance publique en matière de contrôle des licences de transport pour les utilisateurs de deux-roues motorisés. Je n'ai reçu aucune réponse, sûrement parce qu'il n'y a quasiment pas de contrôle : je le sais par les livreurs et par ceux qui travaillent à vélo. Plus précisément, je vous invite à consulter les travaux de la chercheuse Laetitia Dablanc du laboratoire Ville Mobilité Transport, qui vient de nous fournir de nouveaux éléments de mesure : près de 37 % des livreurs utilisent des deux-roues motorisés

connaître leur situation légale, mais cela pose bien des questions. Dernier point : le mythe selon lequel ces travailleurs ne voudraient pas être salariés.

comme l'a dit M. Gay. En effet, la proposition de loi prévoit que, à l'exclusion de ceux qui exercent une activité de transport de personnes, la rémunération des travailleurs des plateformes numériques « devra être constituée sur une base horaire. Suivant sa logique, l'article 1 renvoie à la négociation collective les modes de calcul de tous les éléments de rémunération sans référence à un socle législatif. Les auteurs de l'amendement proposent de fixer, en faisant référence au SMIC,

Je précise aussi que ce dispositif n'est pas incantatoire : il a un fondement juridique qui le rendrait opposable. Examinez-le en détail, on ne pourra pas accuser un donneur d'ordre

à identifier et prévenir les risques d'atteintes graves envers les droits et libertés des travailleurs, leur santé, leur sécurité et, d'autre part, à leur garantir une rémunération décente. Les utilisateurs de plateformes à titre professionnel seraient solidairement responsables de ce devoir de vigilance. Cet amendement va dans le sens d'une meilleure protection des travailleurs des plateformes, mais n'est pas compatible avec ma position, dans la mesure il a pour objet de maintenir les travailleurs concernés dans un statut d'indépendance qui ne peut être que trompeur. Au contraire, le groupe auquel j'appartiens souhaite étendre aux travailleurs concernés les protections du salariat, notamment une rémunération au moins égale

et que la plateforme devrait réparer les dommages occasionnés. Je comprends l'esprit de cet amendement : ce dispositif s'inspire de la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, qui impose aux grandes entreprises et grands groupes d'établir et de mettre en oeuvre un plan de vigilance destiné à identifier et à prévenir les risques d'atteintes graves

en compte dans les directives européennes. Toutefois, en l'espèce, le dispositif proposé ne s'articule autour d'aucun seuil, crée des contraintes qui seraient difficilement vérifiables. il ne nous paraît pas suffisamment abouti pour permettre de respecter des dispositions légales qui seraient, dans certains cas, disproportionnées ou très difficilement applicables. Par ailleurs, ainsi que je l'ai déjà indiqué plusieurs

côté, il y a donc le sujet de la protection sociale des travailleurs des plateformes et, de l'autre, celui des possibilités d'évolution. Toute la philosophie de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel repose sur l'idée qu'il faut permettre l'émancipation professionnelle par le travail et la formation tout au long de la vie.

Carrefour, par exemple, a annoncé pendant le confinement un partenariat avec Uber Eats pour la livraison de ses clients à domicile, ce service étant presque présenté comme un service public. De même, la SNCF développe sous marque blanche un système de réservation préalable de VTC, tandis

l'article 1 A du projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, ma collègue Mireille Jouve souhaitait voter pour.

encore plus prégnante en ces circonstances. En effet, alors que notre pays traverse une grave pandémie, que la baisse d'activité liée au confinement va se traduire très directement par des difficultés accrues pour nos concitoyens, il nous a semblé utile d'assurer un soutien solide aux ménages concernant un poste de dépenses très lourd dans leur budget : les charges de loyer. Malgré les dispositifs de chômage partiel mis en place, de nombreux allocataires des aides au logement affrontent une baisse, voire une suppression de leur revenu. Le confinement a représenté une charge financière supplémentaire : hausse des dépenses alimentaires, utilisation plus importante d'eau et d'électricité, notamment. Selon une note de l'Institut de recherches économiques et sociales (IRES), plus de 2,5 millions de ménages de locataires ou d'accédants à la propriété, soit un tiers des actifs, ont été touchés. C'est considérable. Face à cette situation inédite, le Gouvernement a commencé à agir : report de la trêve hivernale à la fin de l'état d'urgence sanitaire, mise en place d'une aide aux ménages attributaires des minima sociaux, ainsi qu'une hausse de l'aide personnalisée au logement de 100 euros par enfant. Ces actions ponctuelles sont nécessaires, mais insuffisantes sur le long terme. Nous soutenons ainsi les propositions formulées par les associations de création d'un fonds spécifique pour aider durablement les locataires. Pour autant, et sur un temps plus long, il nous semble utile- c'est ce que nous souhaitons engager avec ce texte -de revenir sur toutes les décisions prises qui ont conduit à raboter les aides au logement. L'adoption de cette proposition de loi dès le stade de son examen en commission- j'en remercie mes collègues, ainsi que Mme la rapporteur -envoie un signe clair du Sénat, un signal transpartisan, constructif et positif en faveur d'une priorité donnée à la préservation des aides au logement, qui sont un outil majeur d'égalité et de solidarité pour nos concitoyens. Trop d'économies ont été réalisées sur ce poste de dépenses, pourtant vital pour nombre de familles. Alors que la question du logement est aujourd'hui fondatrice et structurante, le Gouvernement a fait le choix depuis le début du quinquennat de la considérer uniquement comme un produit marchand, asséchant par là même tous les amortisseurs de crise que sont les aides à la personne et les aides à la pierre. Un choix très « ancien monde », si vous me permettez l'expression, monsieur le ministre, l'aboutissement d'une logique libérale appliquée à un bien essentiel. L'habitat est une question politique majeure. Le confinement l'a démontré avec acuité : le logement est l'une des cellules de base indispensables à l'individu. De sa qualité, de sa taille, de sa configuration dans son environnement, de sa proximité avec les services publics dépendront pour beaucoup la qualité de vie de ses occupants, leur capacité à faire société. Le droit au logement est consubstantiel à la notion même de dignité humaine et il est reconnu comme un droit à valeur constitutionnelle, garanti par les textes fondamentaux de la République et considéré comme tel par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Nous ne pouvons donc accepter cette politique du rabot qui a frappé ces aides directes à la solvabilisation des ménages, aides qui bénéficient pourtant à 6,5 millions de personnes.

Cette mesure est apparue particulièrement injuste au moment même où était supprimé l'impôt sur la fortune : 32 millions d'euros économisés sur les Français les plus fragiles et 3,2 milliards d'euros redonnés à ceux qui possèdent déjà tout À ce titre, la crise que nous traversons a permis de revoir cette échelle de valeurs, afin de définir qui sont réellement les premiers de cordée dans notre pays. Ce retour à l'intérêt commun doit nous conduire en cohérence aujourd'hui à effectuer d'autres choix budgétaires, notamment en faveur des employés et des ouvriers, qui représentent 70 % des bénéficiaires des APL : supprimer les niches fiscales inutiles et remettre l'argent là où il est utile pour soutenir le mouvement HLM, permettant ainsi de disposer de logements abordables et d'épauler nos concitoyens pour garantir le maintien dans le logement et l'accès à ce droit essentiel. L'émoi suscité par cette mesure a conduit à la création du collectif Vive l'APL, rassemblant plus de 70 organisations de défense des locataires et mal-logés, d'étudiants, de syndicats et de bailleurs sociaux réclamant le retrait de celle-ci. Depuis a également été créé le Collectif des associations unies regroupant de nombreuses associations oeuvrant dans le secteur social, qui demande notamment de renoncer à toutes les économies réalisées depuis 2017 sur ces aides. Pourtant, le Président de la République s'obstine encore à justifier la réduction de cette aide fondamentale pour nombre de familles, avec un mépris coutumier pour « les gens qui pensent que [ ...] le summum de la lutte, c'est les 50 euros d'APL » et qui ont tant besoin « du pognon de dingue » des aides sociales. Il affirmait aussi ne plus vouloir qu'aucune personne ne soit demain à la rue. Une stratégie du « en même temps » qui ne convainc pas. Cette défense des APL n'est pas une lubie ou un totem c'est la reconnaissance de leur utilité, de leur capacité à jouer les amortisseurs de crise. Il s'agit en effet de l'un des principaux instruments anti-pauvreté dans notre pays. Ce gouvernement, plus que tous les autres, n'a eu de cesse de les attaquer. note un désengagement de l'État de l'ordre de 7 milliards d'euros sur les aides au logement depuis le début du quinquennat. L'ensemble des politiques publiques du logement ont été largement malmenées : extinction progressive des aides à la pierre financées par l'État, disparition de l'aide aux maires bâtisseurs, mise à mal du modèle social des bailleurs HLM, notamment par l'instauration de la réduction de loyer de solidarité, baisse des APL en 2017, absence de revalorisation en 2018, et, enfin, revalorisation en deçà de l'inflation pour 2019 et 2020. Parallèlement, l'APL accession a été supprimée. Dans le cadre de la loi de finances pour 2020, le niveau de revalorisation des APL a également été limité à 0,3 %, en deçà de l'inflation et de l'indice de référence des loyers Selon la réforme engagée par la loi de finances pour 2019 et par la loi de financement de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement doivent faire l'objet d'une réforme de leur mode de calcul liée à la contemporanéité de la prise en compte des ressources. D'après les chiffres dont nous disposons, cette réforme pourrait pourrait entraîner une baisse du montant de ces aides pour 1,2 million d'allocataires, en particulier des jeunes actifs, sur un total de 6,5 millions de bénéficiaires. Et 600 000 allocataires verraient leur prestation purement et simplement supprimée.

Nous proposons donc par le biais du présent texte de changer le curseur et de remettre au coeur de la définition des aides au logement l'intérêt des allocataires. D'autres mesures du domaine réglementaire doivent d'ailleurs être engagées par le Gouvernement, notamment concernant la réforme de la contemporanéité ou la suppression de la baisse de 5 euros, sur laquelle il faudrait revenir. De manière précise, et parce qu'ici nous faisons la loi, nous demandons, par l'article 1de cette proposition proposition de loi, la suppression du délai de carence d'un mois pour le versement des aides personnelles au logement. À l'heure où la crise risque d'accroître le nombre de nouveaux allocataires, il convient en effet de ne pas par l'instauration d'un mois de carence, des difficultés aux difficultés, risquant d'entraîner des familles dans la spirale des dettes locatives et des expulsions locatives. Par l'article 2, nous demandons la suppression de l'application d'un seuil de non-versement, aujourd'hui fixé à 10 euros. Nous avons conscience des réserves sur cet article et nous y reviendrons au cours du débat. L'article 3 initialement proposé visait à créer une présomption de bonne foi lorsque la baisse des ressources est liée à la crise sanitaire pour le maintien des APL. Il a été supprimé en commission au motif qu'il était redondant avec le droit existant. Nous partageons cet avis et en prenons acte. L'article 4 permet, quant à lui, de revenir sur la désindexation des APL opérée par l'article 200 du projet de loi de finances pour 2020. Comme en 2019, celles-ci ne sont revalorisées que de 0,3 % en 2020

Mes chers collègues, nous remercions la commission de nous avoir suivis en adoptant cette proposition de loi. Nous espérons maintenant que la séance sera l'occasion de mener ce beau débat sur les conditions d'un droit fondamental pour nos concitoyens, celui d'avoir un toit, et de ses modalités de mise en oeuvre, qui passent par un soutien aux aides personnelles

La lutte contre le logement cher et le mal-logement doit ainsi devenir prioritaire par rapport aux économies de bout de chandelle réalisées sur le dos d'un trop grand nombre de nos concitoyens, et, parmi eux, de tous ceux qui ont été le plus souvent en première ligne lors de cette crise sanitaire. La parole

aux deux mesures principales de cette proposition de loi visant à garantir l'efficacité des aides personnelles au logement : la suppression du mois de carence et la réindexation des APL sur l'indice de référence des loyers. Nous sommes- à une large majorité

En effet, en 2017, le Gouvernement a décidé, de manière délibérée et brutale, de réaliser des économies sur les aides au logement pour réduire le déficit budgétaire et permettre à la France de sortir de la procédure pour déficit excessif. votre collègue Gérald Darmanin l'a écrit noir sur blanc dans sa réponse aux observations que la Cour des comptes formule dans son rapport public annuel pour 2020. Entre 2017 et 2020, compte tenu de la non-application de la contemporanéisation des APL pour le pour le moment, près de 6 milliards d'euros seront économisés. Dit autrement, entre le budget de 2017 et le budget de 2020, l'État dépense 3 milliards d'euros de moins pour les APL. Or, dans ce même rapport public, la Cour des comptes souligne combien cette politique de baisse uniforme des APL, quelle que soit la situation du foyer, suscite des interrogations en termes d'équité. Elle relève aussi qu'elle a mis à mal la confiance entre le Gouvernement et le mouvement HLM et nui à la capacité des acteurs de se projeter dans l'avenir. Rappelons quelques données. Les APL représentent près de 40 % des moyens financiers de la politique du logement, soit environ 17 milliards d'euros en 2018 et en 2019. De fait, 20 % des ménages français- les plus fragiles -touchent les APL, soit 6,6 millions. Les APL sont l'une des principales mesures de redistribution en leur faveur. Elles représentent un tiers de l'effort de la Nation pour les ménages du premier décile de niveau de vie, qui constituent 75 % des bénéficiaires. Baisser les APL ou ne pas les revaloriser correctement, comme l'a fait le Gouvernement, c'est frapper le portefeuille et le pouvoir d'achat des moins favorisés. C'est aussi accroître les inégalités en réduisant la redistribution. Cette politique de réduction des aides au logement est également- nous le constatons -une politique d'affaiblissement du logement social. La réduction de loyer de solidarité (RLS) qui a été imposée représente une ponction de 1,3 milliard d'euros en 2020. L'ensemble des opérateurs ont été durablement déstabilisés. La capacité des bailleurs à investir, c'est-à-dire à construire de nouveaux logements, a été amputée. D'ailleurs, dans la crise que nous traversons, c'est moins de trésorerie que de fonds propres que vont manquer les bailleurs sociaux. Monsieur le ministre, notre pays va devoir affronter une crise du logement très importante puisque ce sont sans doute près de 100 000 constructions qui ne seront pas réalisées cette année en raison de l'arrêt des chantiers pendant le confinement. Ne serait-il pas temps de se rendre compte que les économies effectuées ces dernières années sont aujourd'hui un handicap pour organiser la relance et soutenir les locataires en difficulté ? En 2008 et en 2009, les bailleurs sociaux avaient pu acheter un grand nombre de programmes en vente en l'état futur

de créer un fonds d'aide à la quittance doté de 200 millions d'euros. C'est moitié moins que l'économie réalisée chaque année par la réduction de 5 euros des APL, moins que leur gel en 2018, moins que leur non-revalorisation en 2019 et en 2020. Pour ma part, comme je l'ai dit à plusieurs reprises à cette tribune, je suis convaincue qu'il faut redonner de l'air aux bailleurs sociaux. La question d'un moratoire de la RLS ou d'une mesure équivalente doit être envisagée. Je crois également à la nécessité du rétablissement de l'APL accession, qui est une mesure peu coûteuse peu coûteuse et efficace pour soutenir l'accession sociale à la propriété. Peut-être nous indiquerez-vous, monsieur le ministre, les intentions du Gouvernement dans le cadre du futur plan de relance. Mes chers collègues, après avoir rappelé les motivations de fond de la commission en faveur d'une

La commission vous propose, tout d'abord, de supprimer le mois de carence de versement des APL lors de leur première demande. Il convient de rappeler que ce mois de carence est plus une mesure budgétaire qu'une mesure Il a été instauré par la loi de finances pour 1995, sachant qu'il s'applique aux prestations familiales depuis 1983. Mais, en réalité, il existe déjà de nombreuses exceptions. Il ne s'applique qu'aux premières demandes, pour le premier mois d'ouverture des droits, et non si les droits sont acquis depuis plus longtemps, mais n'ont pas fait l'objet d'une requête. Par ailleurs, il ne s'applique pas aux personnes hébergées qui accèdent à un logement, à celles qui quittent un logement frappé d'insalubrité, à celles qui sont logées en foyer- jeunes travailleurs et travailleurs migrants -et aux bénéficiaires des minima sociaux. Vos services, monsieur le ministre, nous ont indiqué que le coût de cette mesure serait de l'ordre de 250 millions d'euros en année pleine, 1,2 million de nouvelles demandes étant enregistrées chaque année. J'estime cependant

au détriment des populations les plus fragiles qui bénéficient des APL ; enfin, que, dans le contexte actuel où il est malheureusement à craindre que de nombreux Français ne deviennent éligibles à cette aide, il serait alors incompréhensible de réaliser une économie à leur détriment. La commission vous propose d'approuver une seconde disposition, prévue à l'article 4 de la proposition de loi : le retour à l'indexation des APL sur l'IRL. Comme je l'ai rappelé, après avoir réduit les APL de 5 euros à l'été 2017, le Gouvernement a pris des mesures plus discrètes conduisant à leur érosion par rapport à l'inflation

c'est-à-dire de se baser sur l'IRL, qui aurait conduit à une hausse de l'ordre de 1,5 %, mesure dont le coût aurait été de 171 millions d'euros selon les chiffres qui m'ont été communiqués. d'une demande forte des associations de locataires et de l'ensemble du monde HLM. Nous la soutenons, estimant qu'il s'agit d'une mesure de justice. En revanche, la commission, dans sa majorité, n'approuve pas la suppression du seuil de non-versement, qui est actuellement fixé à 10 euros par mois. L'argument selon lequel le vrai seuil devrait être celui de l'éligibilité et non un montant minimal de versement est naturellement compréhensible, mais il s'agit en l'espèce d'une mesure de bonne gestion. Ce seuil touche actuellement 17 000 ménages pour un montant total de 1 million d'euros et des APL moyennes de 60 euros par an, alors que le coût de gestion et d'instruction d'une demande serait de l'ordre de 80 à 90 euros selon la Cour des comptes. Par ailleurs, il faut le rappeler, en 2017 et en 2018, pour atténuer les effets indésirables de la baisse de 5 euros des APL, ce seuil avait été abaissé de 15 à 10 euros, voire complètement supprimé lorsque la RLS

amendement de suppression de l'article 2. En résumé, la commission souhaite promouvoir une politique du logement juste et ambitieuse, tenant compte des difficultés des locataires, tant dans le parc social que dans le parc privé, et des bailleurs dans le cadre de la crise sanitaire et économique que traverse actuellement notre pays. C'est pourquoi elle vous propose de supprimer le mois de carence et de revenir à une meilleure revalorisation des APL. La parole

a montré à quel point l'habitat est une question cruciale, centrale, malheureusement encore beaucoup trop vectrice d'inégalités sociales. C'est aussi, comme vous l'avez mentionné, madame la sénatrice, une question de dignité pour beaucoup de nos concitoyens.

pour lesquels Mme la rapporteure est extrêmement engagée avec d'autres représentants du monde HLM. Les titres participatifs représentent aujourd'hui près de 900 millions d'euros. L'un des représentants d'une famille d'office d'HLM, pour ne pas le cacher, me disait encore dernièrement au téléphone : si nous avions voulu

Songez qu'hier soir, madame la sénatrice, 180 000 personnes- je dis bien 180 000 personnes ! -ont été accueillies dans les dispositifs de mise à l'abri. Pendant la période de confinement, nous avons ouvert 22 000 places supplémentaires qui permettent d'atteindre ces 180 000 places en réquisitionnant, notamment, bon nombre de chambres d'hôtel.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd'hui comporte des mesures visant à améliorer le régime des aides au logement. Ces dispositions sont importantes, car elles sont porteuses de justice sociale et d'équité. Elles sont d'autant plus nécessaires qu'elles interviennent dans un contexte de début de crise économique et sociale. La pandémie et les mesures prises pour l'endiguer ont eu de graves effets sur notre économie, mais aussi sur celles de nos voisins et partenaires économiques. L'économie française va faire face à une récession jugée historique par le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Avec une contraction de 11 % du PIB en 2020, ainsi qu'un déficit public d'au moins 9 % et une dette publique aux alentours de 115 la crise économique qui est devant nous aura malheureusement des conséquences fortes sur les ménages. Or le logement demeure l'un des premiers postes de dépenses des Français. C'est donc notamment dans ce domaine qu'il faut apporter un soutien aux plus fragiles de nos concitoyens. Au-delà de son caractère social, la politique du logement est également un outil majeur de relance économique. économique. Elle apporte un soutien actif au secteur du bâtiment et à de nombreux corps de métier. Certains bailleurs sociaux qui maillent nos territoires sont déjà très vulnérables ; ils le seront encore davantage en cas de crise. Ils sont des acteurs importants de l'aménagement de nos territoires. Il faut donc soutenir leur capacité d'intervention, d'investissement et de rénovation. Les aides au logement sont un pilier ancien et essentiel de la politique sociale française. Elles sont inscrites dans le paysage français depuis 1948. En 2018, ce sont 17 milliards d'euros qui étaient versés à un peu plus de 6 millions de bénéficiaires. Il importe donc de ne pas faire de petites économies sur les aides sociales au logement, car elles sont souvent lourdes de conséquences. La proposition de loi que nous examinons comportait deux mesures qui ont été supprimées en commission. Il s'agissait, en premier lieu, de la suppression du seuil de non-versement de l'APL fixé à 10 euros. Même si j'approuve son objectif, qui est à première vue louable, cette disposition doit toutefois être confrontée à un principe de réalité et de bonne gestion des fonds publics, notamment au regard du coût

La commission a heureusement supprimé cette disposition, qui vidait de sa substance le principe même d'une aide au logement. Si le loyer n'est pas payé, comment pourrait-on justifier le versement d'une telle aide, qui vise à couvrir partiellement le paiement le paiement du loyer ? Je suis conscient de la nécessité d'appréhender les difficultés de paiement des loyers pour certains foyers en ces temps à venir, mais une telle mesure

si l'aide est due, elle doit être payée dès que les conditions sont remplies. C'est là aussi une question de justice et d'équité. Je suis également favorable au rétablissement de l'indexation de l'APL sur l'indice de révision des loyers. Pour garder toute son efficacité, le montant de cette aide doit être réactualisé régulièrement. C'est là aussi un enjeu d'équité, car cette non-indexation conduit inexorablement à voir s'éroder le montant relatif de l'APL, alors même que les loyers, eux, peuvent faire l'objet d'une indexation. Nous avons fait face ensemble à la crise sanitaire. Pour tenir face à la crise économique, nous avons besoin de soutenir les entreprises, bien évidemment, mais aussi les ménages, car ils sont ils sont un des moteurs importants de la consommation et donc de la croissance. Dans ce sens, l'APL accession était un dispositif utile dont je regrette la disparition. Il permettait aux ménages les plus modestes d'accéder plus facilement à la propriété. Les différentes composantes de notre société sont interdépendantes ; il importe de n'en négliger aucune. Cette proposition de loi ne suffira pas à régler toutes les difficultés, mais elle contribuera utilement à préserver la situation des plus fragiles de nos concitoyens et permettra un certain nombre d'ajustements du dispositif des aides au logement. Nous voterons donc le texte tel qu'il a été amendé par la commission et sur proposition de Mme la rapporteure.

Le logement, et encore plus le logement pour les plus modestes, doit constituer une préoccupation de chaque instant pour les responsables politiques que nous sommes,

La période de confinement que nous venons de traverser nous a démontré, une fois de plus, si c'était nécessaire, à quel point le logement, d'une part, pouvait être source d'inégalités sociales et, d'autre part, constituait un élément essentiel du bien-vivre, voire peut-être demain du bien-travailler. Je l'ai rappelé en commission, sans logement, on ne peut construire sa vie, sa famille, son travail, sa santé. C'est le coeur, le nid, comme le dit Jean-Louis Borloo Différentes problématiques me semblent essentielles à aborder dans nos réflexions actuelles et à venir. Tout d'abord, le rôle des offices d'HLM dans la création et l'amélioration du logement pour les ménages les plus en difficulté est essentiel. Malheureusement, les précédents projets de loi de finances, comme l'a rappelé la rapporteur, et certaines mesures de la loi ÉLAN produisent les effets attendus. Beaucoup d'organismes peinent aujourd'hui à construire et à rénover leur parc de logements sociaux. L'impact de la RLS, concomitante à la diminution de la contribution de l'État aux APL de 3 milliards d'euros depuis trois ans, a contribué tout autant à remettre en cause le modèle économique des bailleurs sociaux qu'à fragiliser certains ménages en difficulté. Cette équation budgétaire imposée complique fortement l'atteinte des objectifs assignés au secteur du logement social, qu'il s'agisse de l'engagement de poursuivre la construction neuve ou de l'accroissement de 25 % des rénovations. La vente d'appartements n'est évidemment pas au rendez-vous pour créer de la trésorerie ainsi que vous l'aviez imaginé. On peut craindre que la crise, qui ne fait que commencer, n'améliore pas la situation. situation. Par ailleurs, comme je l'avais souligné précédemment, on peut légitimement s'interroger sur l'intérêt de vendre des logements locatifs sociaux pour construire d'autres logements locatifs sociaux quand on sait que ce ne sont que très rarement les occupants qui les achètent La crise sanitaire dérive aujourd'hui en crise économique et dérivera demain en crise sociale. Cette situation signifie que nous devons protéger et aider ceux qui vont le plus souffrir. Je le rappelais, les questions de logement constituent l'un des principaux freins au retour à l'emploi. La nécessité de construire plus et mieux, partout en France, est donc importante. Cela doit se faire aussi dans le cadre d'une politique de la ville transversale et puissante. Les ruptures sociales se creusent toujours en période de crise. Nous devrons faire attention et les anticiper.

au 31 décembre 2024, qui risque de ne pas pouvoir être respectée par les collectivités. C'est un sujet qu'il faudra examiner de près. Le problème de la construction de logements est lié aussi aux questions d'investissement d'investissement public : 70 % de l'investissement public est réalisé par les collectivités locales. Ces dernières sont donc un maillon essentiel de la commande publique et de la reprise économique dans les territoires, en particulier pour les entreprises du bâtiment. Elles ont aussi un rôle à jouer dans la construction et la rénovation de logements. Soyez vigilant à ne pas couper les capacités d'investissement des collectivités, comme vous l'avez fait pour les bailleurs sociaux dans le cadre de choix budgétaires. Votre gouvernement appelle à faire confiance aux maires en cette période de déconfinement progressif. Étendez cette volonté à l'investissement local et aux autres élus locaux. Établissez des relations claires et franches avec tous les niveaux de collectivités. Là encore, j'appelais largement à une telle concertation lors des débats sur la loi ÉLAN. Vos réformes étaient sans doute calibrées pour des moments où l'on navigue par beau temps. Quand la tempête est là, comme aujourd'hui, elles ne permettent pas d'amortir le choc et de maintenir le cap. Bien au contraire, elles pourraient accentuer les difficultés sociales et compliquer encore davantage l'équation du secteur du logement social. Il faudra donc, monsieur le ministre, comme le rappelait Mme la rapporteur, engager rapidement et en premier lieu le moratoire de la RLS tant attendu par les bailleurs sociaux.

Comme j'ai pu le souligner lors de l'examen de la proposition de loi en commission, ce texte vient à point nommé. Même s'il ne résoudra pas tous les problèmes du monde du logement en général et du logement social en particulier, même s'il n'aidera pas toutes les personnes qui ont des difficultés en fin de mois pour régler leur loyer et leurs charges, il va néanmoins dans le bon sens. Il traite des difficultés réelles et apporte, à son échelle, un peu d'oxygène aux ménages. Cet oxygène, le Gouvernement a senti qu'il était nécessaire quand il a décidé d'allouer une prime de 150 euros aux ménages les plus modestes qui percevaient le revenu de solidarité active (RSA) ou par enfant pour les mêmes ménages et pour ceux qui perçoivent l'APL. Par ce mécanisme, vous reconnaissez indirectement, monsieur le ministre, que les minima sociaux et les aides publiques aux ménages ne suffisent pas durant cette période de crise sanitaire, mais aussi, sans doute, le reste du temps. La proposition de loi de mes collègues du groupe CRCE peut vous permettre d'y réfléchir plus précisément. Elle contient des mesures de bon sens que nous soutenons. La suppression du mois de carence dans la perception des APL est une mesure de justice. À l'heure où le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est devenu possible et se justifie par sa contemporanéité, à l'heure où les APL, comme vous le souhaitez, sont versées en prenant en en prenant en compte la situation réelle et immédiate des revenus des foyers, il nous semble logique de ne plus pénaliser les ménages par ce mois d'attente. De même, la réindexation du montant des APL sur l'indice de référence des loyers permettra de suivre la réalité des évolutions économiques du pays. Elle suit la même logique : à situation donnée à l'instant doit correspondre une aide juste et équivalente à ce même instant. Concernant les autres articles, nous soutiendrons les positions de la commission et de Mme la rapporteur, je pense en particulier à l'amendement de suppression de l'article 2 sur le seuil de non-versement. Pour conclure, je me réjouis que la commission ait toujours veillé à ces questions liées au logement et défendu des positions communes, qui vont bien au-delà de nos différences quand il s'agit de financer nos politiques de logements sociaux et nos ménages les plus modestes. La situation actuelle le justifie, ainsi que celle à venir. Vous l'aurez donc compris, les sénatrices et sénateurs du groupe Union Centriste voteront en faveur de ce texte, tel qu'il ressortira de nos débats. La parole

Il faut sans doute beaucoup plus anticiper et aider les plus fragiles à traverser la crise. L'augmentation du chômage nécessite des mesures fortes pour empêcher de nombreux Français de basculer dans la précarité. Il y a urgence pour leur permettre c'est l'objet du texte que nous examinons aujourd'hui -tant dans le parc public que dans le parc privé pour lequel nous avons aussi beaucoup d'inquiétudes. Les aides personnelles au logement représentent plus de 40 % de l'effort public pour le logement. Elles réduisent la charge de logement de 7 millions de ménages locataires bénéficiaires. Or ces ménages ont subi des baisses de revenus du fait notamment du chômage partiel et de l'arrêt de travail pour de nombreuses professions. Quand on a 1 500 euros de revenus avec deux enfants et un reste à charge de 300 euros, c'est très difficile. Il n'y a qu'à voir comment la baisse de 5 euros des APL a été perçue ! Le montant des aides au logement est donc non seulement indispensable pour les soutenir, mais il ne suffira pas pour de nombreux ménages. Il faut aller plus loin et prévoir sans doute pour une période temporaire de nouvelles mesures d'aide qui permettront aux plus fragiles de surmonter leurs difficultés. Il va falloir, là aussi, faire jouer la solidarité nationale, comme beaucoup d'associations le demandent. La crise sanitaire que nous traversons se double d'une crise économique et sociale. Le Gouvernement vient malheureusement d'annoncer une récession de plus de 11 %.

dans la protection des personnes. Cette urgence sociale est relayée depuis des semaines par les acteurs de la solidarité que nous avons beaucoup auditionnés avec Mme Estrosi Sassone, mais également par les bailleurs sociaux et les associations d'élus. (FSL) est particulièrement mobilisé pour venir en aide aux ménages fragilisés, mais les locataires ayant des difficultés à payer leur loyer qui ne sont pas éligibles à ce fonds ne disposent pas d'aide spécifique. Le FSL n'est d'ailleurs pas universel puisqu'il est destiné aux personnes en grande situation de précarité sociale et est attribué selon des critères propres à chaque département.

eu et ont encore des effets irrémédiables qui installent une crise durable de la construction de logements abordables, de la réhabilitation et de la rénovation urbaine, dont les effets seront encore amplifiés par La France doit produire du logement abordable- or, nous le savons, il y aura environ 100 000 logements en moins -et soutenir les familles modestes. Comment résorber l'habitat indigne si l'on ne peut pas reloger les familles ? Comment mettre en place la politique dite du « logement d'abord » sans offre de logements adaptée et sans financement de l'accompagnement social ? Comment demander aux maires de mettre en oeuvre des politiques publiques quand ils n'en ont plus les moyens ? Comment donner confiance à notre jeunesse lorsque la précarité s'installe et que le logement devient inaccessible ? S'agissant des aides au logement, les décisions successives du Gouvernement durant ces trois dernières années ne sont pas allées dans le bon sens : baisse de 5 euros des APL, gel de leur barème en 2018 et sous-indexation à hauteur de 0,3 % en 2019 et 2020-

78 milliards de rentrées fiscales. Il ne faut pas l'oublier ! Le logement doit cesser d'être la variable d'ajustement du budget de l'État, même si vous nous assurez que vos choix politiques ne sont pas purement budgétaires.

deçà des plafonds de ressources. Il est donc urgent de réorienter la politique du logement, et la question des aides au logement en est l'illustration la plus édifiante. Par

Après avoir favorisé le chômage partiel, la dépense publique ne parviendra pas, malheureusement, à sauver toutes les entreprises qui annonceront leur faillite et les emplois correspondants. À défaut de revenu universel, les aides sociales constituent un soutien précieux permettant à nos concitoyens d'amortir le choc provoqué par une diminution ou une perte totale de revenus qui risque de compromettre, en particulier lorsqu'ils sont locataires, Des moyens supplémentaires doivent être pensés pour permettre le maintien dans leur logement actuel, avant que ne s'enclenche l'engrenage de la précarité. Nombreuses sont les associations qui nous alertent sur ce point. Certes, la vague des impayés n'est pas encore arrivée. Pour autant, elle ne saurait être prématurément écartée. Il est donc fortement souhaitable de l'anticiper et d'éviter les expulsions en cascade.

Si le prolongement de la trêve hivernale jusqu'au 10 juillet constituait une impérieuse nécessité, je regrette l'absence d'initiative de l'État sur le long terme au profit des locataires, en ces temps incertains marqués par une réelle

CLCV constate des abus. Les aides personnelles au logement sont des aides sociales ; elles ne doivent pas servir à financer les surtarifications de loyers. Aussi, même si elle ne peut tout résoudre au regard des limites de l'initiative parlementaire, la présente proposition de loi prévoit des aménagements en matière de modalités de versement et de détermination du montant des APL que l'on ne peut que soutenir. Les deux principales mesures proposées auront un effet positif perceptible pour les ménages. Tout d'abord, la suppression du mois de carence paraît plus que pertinente, car elle contribuera au paiement du premier loyer des personnes nouvellement éligibles aux APL. Ce n'est pas sans intérêt, au vu de la forte probabilité d'une augmentation des demandeurs dans les mois à venir. De même, la réindexation des APL sur l'indice de référence des loyers soit une revalorisation d'environ 1,5 % au lieu de 0,3 %, est socialement juste et cohérente du fait de l'évolution du poids de la dépense de logement sur les budgets des ménages. En revanche, nous sommes partagés sur la suppression du seuil minimal de non-versement des APL, qui trouve sa justification dans la couverture des coûts de gestion. Des montants aussi faibles d'APL, en deçà de 10 euros, sont incompréhensibles, y compris pour les bénéficiaires.

La proposition de loi vise ainsi à renforcer l'efficacité des APL. Elle évoque un débat ancien qui subodorait l'existence d'un potentiel effet inflationniste : le risque de la prise en compte par le bailleur du montant de l'allocation dans la fixation du loyer, notamment en période de pénurie de logements. Or cette pénurie est structurelle dans les zones tendues, et le choc de l'offre n'a pas encore eu lieu. Si un effet inflationniste est démontré, la réalisation d'économies sur les APL de manière uniforme pénalise cruellement les ménages victimes des défaillances d'un marché aux équilibres fragiles. L'optimisation de l'intervention publique dans le domaine du logement est souhaitable, mais elle ne doit pas manquer son objectif premier, qui est avant tout social. Parmi ces ménages, nous ne retrouvons pas uniquement ceux qui subissent des accidents de la vie. Dans les zones tendues, les travailleurs percevant un salaire moyen, qui sont souvent ceux qui se sont révélés indispensables au fonctionnement du pays et que tout le monde a remerciés, peinent à payer leur loyer. Je ne reviendrai ni sur le contexte budgétaire ni sur les économies réalisées dans le cadre de la politique du logement au cours de ces dernières années. Les auteurs de la proposition de loi et d'autres intervenants ont pu le rappeler, la donne a changé. Une crise conjoncturelle s'ajoutant à une crise structurelle, il est impératif de se réinventer pour l'avenir. Le télétravail, qui s'est imposé après une longue hésitation des entreprises, apportera peut-être du lest et permettra de rééquilibrer notre territoire, Français ayant pu goûter à des conditions de vie plus sereines en dehors des milieux urbains. Nous espérons que ces changements profonds auront un effet positif sur l'accès au logement. Mais cela ne nous exonère pas de la responsabilité de donner un coup de pouce immédiat aux locataires.

La complexité des critères de versement est telle qu'« une volumineuse plaquette décrivant leur mode de calcul » était éditée jusqu'en 2013. Elle ne l'est plus depuis, fort heureusement. poursuis ma lecture : « Le nombre de paramètres de calcul accentue le risque d'oublis ou d'erreurs, la complexité de ce calcul ne permettant pas de repérer immédiatement une éventuelle incohérence. Simplifier le mode de calcul des aides est désormais indispensable : au-delà des coûts de gestion qu'elle génère,

Cette nouvelle disposition « devrait constituer une réelle avancée. Cela permettra de mieux fiabiliser les montants de ressources pris en considération dans le calcul et d'adapter le niveau de l'aide à la situation réelle du bénéficiaire.

Nos collègues communistes considèrent que la politique menée depuis le début du quinquennat en matière de logement a conduit à une précarisation accrue des ménages à revenus modestes, et ils proposent quatre mesures pour infléchir cette politique : la suppression du délai de carence d'un mois pour le versement des aides personnelles au logement ; l'abrogation du seuil de non-versement des APL, actuellement fixé à 10 euros par mois le maintien des APL en cas d'impayés de loyers dans le cas d'une crise sanitaire ; la réindexation des APL sur l'indice de référence des loyers en 2020. La commission des affaires économiques du Sénat s'est prononcée favorablement sur deux mesures : le délai de carence et la réindexation des APL sur l'indice de référence des loyers. Elle a considéré, à juste titre, que la politique menée jusqu'à présent avait pénalisé les ménages les plus en difficulté et qu'elle risquait d'amplifier ces difficultés au regard de la crise économique catastrophique qui s'annonce, comme l'ont dit plusieurs de mes collègues. Au-delà des Au-delà des mesures proposées par nos collègues communistes et de celles qu'a retenues la commission, se pose la question de la pertinence et de l'efficacité des politiques de logement menées depuis de nombreuses années, singulièrement depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Je salue le travail fourni et constant de ma collègue rapporteur sur ce sujet. Nous voyons bien que la régulation budgétaire, qui sape le pouvoir d'achat des plus modestes et aggrave la précarité des ménages, ne peut tenir lieu de politique. L'enjeu n'est pas mince. Je rappelle que les trois aides personnelles au logement sont versées à 6,6 millions de ménages et permettent une diminution importante de la charge des dépenses de logement des locataires qui en bénéficient. La Cour des comptes relève qu'elles couvrent en moyenne 49 % du loyer hors charges, dans le cas de l'APL versée aux locataires de logements sociaux, et environ 36 % du loyer pour ce qui concerne l'allocation de logement familial et l'allocation de logement social versées aux ménages logés dans le secteur locatif privé. En 2015 et 2017, ces trois aides atteignaient 18 milliards d'euros par an. Elles ont été ramenées à 17 milliards d'euros en 2018 et 2019, et la loi de finances pour 2020 prévoit un montant stabilisé à 15,3 milliards d'euros. Les deux mesures décidées au deuxième semestre de 2017- la réduction uniforme des APL de 5 euros par mois, et la mise en place d'une réduction du loyer de solidarité dans le parc locatif social -n'ont eu d'autre objectif que de réduire le déficit des finances publiques. Elles ont fortement ébranlé l'opinion publique et suscité une vague de contestation. Elles succédaient à de nombreuses mesures de régulation, moins visibles, prises par le gouvernement de François Hollande, comme le gel ou la sous-indexation des paramètres de calcul, la dégressivité de l'aide pour les loyers les plus élevés, la prise en compte du patrimoine des bénéficiaires, ou encore la suppression de l'aide pour les accédants à la propriété. Les évolutions attendues à partir de cette année- je pense, en particulier, à la prise en compte contemporaine des ressources des bénéficiaires pour le calcul des aides, dont la mise en oeuvre a d'ailleurs été repoussée à plusieurs reprises, tant elle est complexe -et le projet de création d'un revenu unique d'activité regroupant l'ensemble des aides à la personne nous laissent craindre une poursuite de cette politique récessive en matière de logement.

Si je ne méconnais pas la nécessité de maîtriser les dépenses, je considère qu'il est temps, monsieur le ministre, de refonder la politique du logement et de remettre l'équité du système au coeur de vos préoccupations. Cette équité, selon la Cour des comptes, passe par l'analyse fine de la situation des personnes disposant de revenus d'activité très modestes, fortement pénalisées en matière d'aide au logement par rapport à celles qui bénéficient de revenus de transfert. Elle passe également par une meilleure information des allocataires potentiels des aides au logement, qui sont environ 2 % à ne pas demander le bénéfice de l'APL la question du non-recours n'est pas sans incidence sur la situation de pauvreté de certains ménages. Une réforme véritablement ambitieuse aurait pour objectif une simplification des règles de calcul des aides. La Cour des comptes regrette, à juste titre, que les pouvoirs publics n'aient toujours pas mis fin à la complexité de ces modes de calcul, à l'origine de nombreux indus et de fraudes. Je ne reviendrai pas sur la perte de confiance des bailleurs sociaux vis-à-vis des pouvoirs publics, survenue à la suite de la réforme du mouvement HLM et de la réduction de loyer de solidarité, décidée unilatéralement. il me semble nécessaire de s'interroger sur les moyens qui doivent être effectivement alloués aux bailleurs sociaux pour relancer l'effort de construction, qui s'avérera indispensable. Je l'évoquais au début de mon intervention, la crise économique s'annonce particulièrement violente, avec un risque de paupérisation d'une partie de la population. Les besoins en logements sociaux, voire très sociaux, seront importants, et la solvabilité des ménages devra être assurée au moyen des aides au logement. Or les objectifs de construction ne seront à l'évidence pas atteints cette année, compte tenu de l'arrêt des chantiers durant la crise sanitaire. La reprise sera lente et allongera les délais de livraison. je souhaite que le Gouvernement soit attentif au rôle essentiel du logement social et des aides personnelles au logement, qui permettent de satisfaire les besoins essentiels des catégories modestes ; un véritable engagement doit être pris à très court terme contre le mal-logement et la précarité, qui fracturent notre société et laissent tant de monde sur le bord du chemin.

Avant le début de la période hivernale, nous étions aux environs de 145 000 ; c'est donc 35 000 places de plus depuis le 1 novembre dernier.

Ce seuil existe pour toutes les prestations, afin d'optimiser le travail des caisses ; 17 000 ménages seraient concernés. Je tiens à rappeler deux choses : c'est ce gouvernement qui, en 2017, a abaissé ce seuil à 10 euros, contre 15 euros depuis 2007

Cet article pose également la question de la charge de travail supplémentaire qui serait alors imposée aux caisses, au vu du nombre de dossiers supplémentaires- on parle tout de même de 17 000 dossiers -et alors que les frais représentés par la liquidation de l'aide dépasseraient le montant de celle-ci. Par conséquent, vous l'aurez compris, le groupe La République En Marche votera pour l'amendement de suppression de la rapporteure, considérant que cette mesure risque de mettre en tension les effectifs des caisses.

à 10 euros, mais c'est aussi lui qui a mis en place la réduction de loyer de solidarité et qui a fait en sorte que le seuil de non-versement n'existe plus dans le parc social, en